a sidéré la Nation tout entière. Oui, en France, si souvent qualifiée de « pays des Lumières », un homme, un enseignant, a été tué sauvagement, parce qu'il transmettait le savoir et la réflexion, parce qu'il transmettait l'humanité pour que ses élèves deviennent demain des femmes et des hommes libres Cette humanité si profonde, qui est au coeur de la laïcité, c'est ce qu'a voulu tuer ce terroriste au nom d'un islam radical. Oui, l'islam doit sortir de l'emprise intégriste encouragée par des pays qu'il faudra dénoncer ! Il faudra aussi permettre, comme ils le souhaitent, à l'immense majorité des musulmans de pratiquer leur religion dans la sérénité. Ce combat devra rejeter les amalgames et les tentatives de récupération et de division qui se multiplient. Samuel Paty est mort en héros. Il a porté au plus haut niveau les valeurs de la laïcité et de la liberté d'expression, jusqu'à en perdre la vie. Son petit garçon pourra être fier de la gloire de son père, en écho à ces hussards de la République, qui, au début du siècle dernier, ont diffusé par l'école publique, partout en France, la nécessité de l'émancipation humaine par le savoir et la culture. Monsieur le Premier ministre, avec la Nation tout entière, nous devons nous lever pour saluer la mémoire de Samuel Paty et entourer ses proches de notre profonde affection, mais nous devons aussi nous lever pour donner enfin aux enseignants les moyens de leur action essentielle pour l'avenir de notre pays. Ces hussards de la République, qu'ils soient à l'école, à l'hôpital, dans les mairies ou les commissariats, sont trop souvent abandonnés. Ils crient ou taisent leur impuissance à remplir leur mission. Il n'y aura pas de réponse à long terme au défi sanglant du terrorisme islamiste sans une véritable reconquête républicaine, qui pose la question clé d'un choix de société plaçant l'humain au coeur des décisions. C'est la voie pour préserver l'unité de la Nation. Avec Gambetta, j'affirme : « Ce qui constitue la vraie démocratie, ce n'est pas de reconnaître des égaux, mais d'en faire. » En ce jour de deuil national, nous nous inclinons devant la dépouille de Samuel Paty, mais nous portons l'espoir que sa mort remettra en mouvement la République laïque, démocratique et sociale, pour que liberté et progrès règnent sur notre territoire. C'est là notre devoir.

une cérémonie d'hommage national à ce professeur lâchement assassiné dans des conditions particulièrement odieuses et inacceptables, de surcroît- vous l'avez rappelé, et

c'est bien la République qui est visée. Au coeur de la République et de ses valeurs figurent évidemment l'éducation nationale, la liberté d'enseigner, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. Telles sont bien, au-delà de la les cibles de cet ennemi que nous connaissons et que nous devons nommer : l'islamisme politique, l'islamisme radical, qui est l'un des terreaux du terrorisme. Les

nous monter les uns contre les autres, d'affaiblir la République, de nous pousser à faire ou à dire des choses qui ramèneraient dans leurs filets encore davantage d'adversaires de la République. Nous agissons de manière ferme et déterminée. Je pourrais évidemment détailler devant la Haute Assemblée les dispositions qui ont été prises

Voyez comme va arriver à point nommé le projet de loi annoncé aux Mureaux voilà quelques jours par le Président de la République pour lutter contre toute forme de séparatisme

Voyez que, dès aujourd'hui, un groupement de fait répandant la haine a été dissous par le conseil des ministres ! Sachez que d'autres suivront.

Mais nous vaincrons. Nous vaincrons dans l'unité et dans la détermination, parce que ces valeurs de la République, nous les partageons. Nous agirons, nous continuerons à agir sans relâche pour que force reste à la loi républicaine. La parole

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale. Toutes nos pensées vont à Samuel Paty, assassiné parce qu'il faisait son métier. Toutes nos pensées vont à sa famille, à ses élèves et à ses collègues, à tous les professeurs qui sont retournés dans leur classe pour accomplir la plus belle des missions qui soit : enseigner, transmettre. Nous le savons, ils y retournent choqués. Ils se sentent parfois trop seuls. Cet attentat terroriste islamiste caractérisé fait suite à d'autres actes barbares animés par la même idéologie. Il y a eu près de 300 morts depuis 2011. Des enfants ont aussi perdu la vie. Face à ce constat tragique, il ne faut pas trembler ; il ne faut pas de compromission. C'est une chose de le dire, mais la question de l'accompagnement au quotidien se pose. En ce moment même, des propagateurs de haine officient encore sur les réseaux. En ce moment même, une lycéenne ne peut toujours pas retourner dans son lycée pour avoir critiqué une religion. C'est inimaginable et inacceptable ! Face à cela, le risque serait de s'autocensurer, de reculer collectivement. Nous parlons là de l'essentiel, des fondements mêmes de notre Nation : la liberté de conscience, le libre examen, la libre expression, l'esprit critique, l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous parlons là de ce que nous sommes : une République laïque, une et indivisible. Nous savons la détermination du Gouvernement et du Président de la République à terrasser cette idéologie mortifère. Le texte sur les séparatismes arrive bientôt au Parlement. Il fera partie de la réponse globale. Monsieur le ministre, comment l'éducation nationale doit-elle accompagner les professeurs dans l'enseignement de la laïcité face à des contestations d'élèves ou de parents violentes jusqu'à l'extrême ? Comment mieux les protéger dans tous leurs enseignements ? de leur formation et de leur encadrement ?

odieusement assassiné par un terroriste islamiste. Un professeur a été assassiné. Ce n'est pas par hasard. L'islamisme politique, cet extrémisme qui ne peut ni ne doit être confondu avec la religion musulmane, celle de bon nombre de nos concitoyens, doublement meurtris aujourd'hui, développe une offensive idéologique obscurantiste contre tout ce qu'incarne la République indivisible, sociale, démocratique et laïque. C'est sur la base de ce qu'il a semé dans les esprits par de multiples réseaux, bénéficiant de nombreuses complaisances ou aveuglements, qu'un terroriste s'est senti encore « autorisé à tuer. Un professeur a été assassiné. Il était de celles et de ceux qui, au quotidien, avaient pour mission de permettre à nos jeunes de devenir des citoyennes et des citoyens émancipés, capables d'exercer leur liberté individuelle de jugement et d'expression, c'est-à-dire de leur permettre d'échapper à des assignations à résidence communautaire, familiale, culturelle, religieuse, sociale ou territoriale. Un professeur a été assassiné. Il était de celles et de ceux qui, dans des conditions souvent difficiles, à contre-courant des haines qui se déversent impunément, devaient expliquer que les femmes et les hommes sont égaux, que personne ne peut être discriminé en raison de son origine, de sa religion, de sa couleur de peau ou de son orientation sexuelle et qu'aucune loi religieuse ne peut s'imposer à la loi de la République. Un professeur a été assassiné. Alors, je vous demande d'affirmer avec force que personne n'est supérieur au professeur de l'école de la République laïque pour la transmission de nos valeurs fondamentales ! Je vous demande aussi d'honorer les 900 000 enseignants, ces piliers de la République, en les protégeant mieux, en renforçant leurs moyens et en les valorisant aux yeux de toute la société ! Ce serait le meilleur hommage à M. le professeur Samuel Paty.

Nos pensées vont bien sûr vers Samuel Paty, à sa famille et à ses proches, à qui nous adressons notre compassion. Elles vont aussi aux forces de l'ordre, qui sont intervenues dans le plus grand professionnalisme.

Assez de minutes de silence, de marches hommages et de reculs ! Notre pays a besoin d'actes forts pour préserver notre démocratie. Car tel est bien l'enjeu du combat culturel qui se nourrit de la misère sociale et dans lequel nous sommes entrés pour au moins Aujourd'hui, l'école, le creuset de l'avenir de notre Nation, a été attaquée. Un enseignant a été décapité pour avoir enseigné la liberté d'expression. Rendons-nous compte du sens terrible de cette phrase J'ai été professeur d'histoire-géographie. J'ai enseigné l'histoire de France à des élèves de toutes origines et de toutes croyances. J'ai tâché de leur transmettre ce qu'a été l'édification de la République par les grands principes émancipateurs des Lumières. J'ai voulu qu'ils apprennent le doute raisonnable, le libre arbitre, le débat contradictoire, afin qu'ils deviennent des citoyens éclairés et d'égale dignité, quel que soit leur milieu d'origine. Mon groupe a toujours été, depuis 1892, un défenseur acharné de la laïcité une laïcité qui ne peut se concevoir que sans adjectif, pour garantir dans la concorde civile l'unité nationale au-delà des opinions et croyances ; une laïcité qui assure le droit de croire ou de ne pas croire, qui permet l'égalité des chances, qui ne réduit pas les individus à une vision essentialiste ; une laïcité à rebours du projet obscurantiste que des fanatiques ne concevant la vie que par le dogme religieux veulent nous imposer. Monsieur le Premier ministre, l'autorité de l'État n'a cessé de reculer depuis trente ans sur la laïcité. Allez-vous enfin mettre un terme à

rendre hommage à nos forces de sécurité intérieure. Dois-je rappeler à la Haute Assemblée que l'auteur de l'attentat, lui aussi barbare, perpétré devant

sauvage de Samuel Paty a été neutralisé par les forces de sécurité quelques minutes seulement après la commission des faits ? Sous

renforcer la laïcité. Cet événement tragique doit nous donner plus fortement encore l'occasion de nous rassembler autour de cette belle valeur

l'éducation nationale. Ma première pensée va à la famille de Samuel Paty, à sa femme et à son fils. La violence de cet assassinat montre l'immense difficulté et la mission essentielle du métier de professeur aujourd'hui. Immense difficulté, car les enseignants sont depuis plusieurs années en première ligne face aux événements tragiques auxquels nos enfants sont confrontés. Mission essentielle, car il s'agit d'accompagner tous les enfants de la République sur le chemin de la connaissance et de la réflexion, gage et moyen d'une vraie liberté de pensée. L'éducation et la construction de l'esprit critique sont les conditions de la démocratie et de la lutte contre le terrorisme. À côté de cette tragédie, combien d'enseignants sont confrontés à d'énormes difficultés dans leur pratique quotidienne ? Les relations se tendent, et l'accompagnement, le soutien et la formation manquent trop souvent cruellement. Nous assistons à une paupérisation du service public de l'enseignement. Cela laisse aujourd'hui les professeurs seuls garants des principes de la République. Il n'y a plus de formation continue digne de ce nom, en particulier s'agissant de la citoyenneté et du vivre ensemble. Pourtant, le besoin est réel. Il faut des dispositions effectives pendant le temps scolaire, avec des moyens de remplacement appropriés. Monsieur le ministre, pour avoir été enseignante en collège pendant trente ans, c'est avec beaucoup d'émotion et d'inquiétude pour l'avenir que je vous demande quel plan de formation ambitieux vous allez mettre en oeuvre dès la rentrée de novembre. Allez-vous proposer un énième numéro vert ou prendre de véritables mesures pour accompagner comme il se doit les professeurs face aux enjeux actuels ? Il est important d'honorer la mémoire de Samuel Paty en poursuivant son travail. La parole

devenu l'écosystème du complotisme, de la haine et, désormais, des influenceurs islamistes. L'assassinat de Samuel Paty a été préparé par les torrents d'injures des fanatiques sur les réseaux antisociaux. Il y a aussi sur ces réseaux ceux qui fracturent méthodiquement notre pays : les identitaires, les racialistes, les indigénistes, les décoloniaux. Il y a enfin les idiots utiles qui crient à l'islamophobie ou au racisme dès qu'on annonce des mesures pour combattre l'islamisme. L'Assemblée nationale a voté la loi qui imposait le retrait des contenus haineux dans les vingt-quatre heures. Cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression, ce qui laisse le problème entier. La liberté d'expression ne consiste pas à mettre en ligne la haine, le harcèlement, les appels au meurtre ou le djihadisme. La loi interdit à la presse de publier de tels contenus, et la presse s'y conforme, sans que personne y voie une atteinte à la liberté d'expression. Les plateformes, quant à elles, s'en exonèrent sans aucune sanction. Les résultats sont sous nos yeux ! Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé hier la création d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui par internet. Pourquoi pas ! Mais il faut aller plus loin. La seule façon de nettoyer le dépotoir des réseaux antisociaux, le « torrent de boue », disait le président Larcher, est l'obligation de retirer les contenus haineux. Il faut absolument y revenir sous une forme acceptable par le Conseil constitutionnel. Nous le devons à Sonia Mabrouk, à Mila,

avec des lois enfin efficaces le cours qu'il donnait à ses élèves, ce cours par lequel il luttait contre la haine et pour l'unité de la République. La parole est à M. le Premier ministre.

et la charia immédiatement exécutée. Mais, cette fois, quelque chose a changé. Les Français sont passés presque instantanément d'un état de sidération à un état de colère ils demandent des comptes, ils exigent des résultats, tout simplement parce qu'ils sentent confusément, mais indéniablement, que nous sommes en train de perdre le combat contre le totalitarisme islamiste.

un combat global contre le désordre migratoire- l'un des terreaux de l'islamisme -, qui est un défi et un obstacle à l'assimilation de nos valeurs républicaines ! Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à êtes-vous prêt à mener ce combat, qui doit être global ? Vous nous parlez d'un texte qui nous arrivera dans cinq mois, en février. Ce texte comportera-t-il, oui ou non, des mesures pour remédier à ce désordre migratoire ?

vous avez dit, à juste titre, que les Français ont été sidérés, qu'ils sont en colère. Je crois que nous le sommes toutes et tous, il n'y a pas de doute là-dessus, mais le Gouvernement de la République que j'ai l'honneur de diriger n'est pas simplement sidéré

Ne désignez pas la France comme une coupable perpétuelle. Ne faites pas comme le Président de la République, qui a déclaré que la France était coupable de crimes contre l'humanité, le pire des crimes ! Monsieur le Premier ministre, il faut réarmer la République et faire aimer la France. Relevons ensemble

Alors, notre pays ne doit pas être faible et nous devons être capables de faire appliquer les décisions judiciaires et administratives. Des milliers d'étrangers qui sont des prêcheurs de haine et veulent abattre les principes de notre République continuent de vivre sur notre sol. Des décisions les ont pourtant condamnés à quitter notre territoire national ; ils sont nombreux, trop nombreux, à être toujours là. Une immense majorité de nos concitoyens, pris d'une colère froide, se pose cette question : pourquoi sont-ils encore là ? À cette question mille fois posée, on nous a mille fois répondu : « Ah oui, mais, vous comprenez, c'est compliqué ... » Où est le ministre de la justice ? Après ce nouvel attentat atroce contre Samuel Paty qui nous a tous touchés très profondément, vous allez être tenté de proposer de nouveau au Parlement de durcir notre arsenal juridique et d'aggraver les peines. En réalité, l'affaiblissement de l'État n'en serait que renforcé, car, le premier problème, c'est l'application ferme et systématique du droit. Or nous savons tous que tel n'est pas le cas. Plus qu'un constat d'impuissance, c'est un terrible aveu. Le Président de la République a annoncé vouloir prendre des mesures concrètes et rapides. Monsieur le ministre de l'intérieur, vous avez indiqué dimanche que 231 étrangers dangereux allaient être expulsés. Pouvez-vous prendre l'engagement de revenir dans un mois nous dire combien d'entre eux sont effectivement partis ? Et pouvez-vous nous donner de la visibilité pour les mois qui viennent ?

Alors, si certaines personnes étrangères condamnées sont toujours sur notre sol dans un mois, il faudra nous expliquer pourquoi. Si ce sont des raisons juridiques, il faudra nous dire précisément lesquelles et modifier la loi. Si ce sont des raisons diplomatiques, il faudra l'expliquer aux Français et prendre toute mesure pour que les obstacles soient levés. J'ai conscience qu'en répondant à ces questions on ne traite qu'une partie du problème. Beaucoup de ces prêcheurs de haine sont Français, comme vous et moi, mais renvoyons déjà en dehors de nos frontières ceux qui méritent de l'être

Paccaud, pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'au garde des sceaux. Si je suis sénateur, je reste le professeur d'histoire-géographie que j'ai été, comme d'autres ici. Vendredi, un enseignant d'histoire-géographie, Samuel Paty, a été sacrifié sur l'autel du fanatisme islamiste, ce fascisme d'aujourd'hui, condamné à devenir martyr pour avoir accompli son devoir- enseigner la tolérance, tenter d'éveiller les consciences -, décapité pour avoir simplement fait son métier, transmis un savoir. L'histoire et sa fille naturelle, l'éducation civique, sont des matières plus que précieuses, parce qu'elles révèlent nos racines, donnent un sens au long fil d'Ariane qui nous relie à nos aïeux, nous permettent de mieux comprendre comment vivre ensemble. Mieux vaut savoir d'où l'on vient pour ne pas se perdre et s'égarer sur les sentiers du malheur, telle est la leçon de vie, le talisman prudent, qu'offrent l'histoire et ses professeurs. Or, depuis des années, ceux qui enseignent l'histoire et l'éducation civique sont parfois menacés. On veut les faire taire La Shoah, les croisades, les valeurs républicaines, la laïcité, les droits de l'homme, la femme égale de l'homme, les islamistes veulent en effacer les traces, ils veulent aveugler les esprits. Et certaines autorités ne veulent surtout pas de vagues- pensez que Samuel Paty avait été convoqué au commissariat pour se justifier Aussi est-il temps de réellement protéger les professeurs et de sanctuariser les cours d'histoire et d'instruction civique, mais aussi ceux de sciences, de lettres ou de sport. Monsieur le ministre, ne doit-on pas désormais instaurer un délit d'entrave à la liberté d'enseigner dans le cadre, bien évidemment, des programmes définis par l'éducation nationale ? C'est l'un des moyens de faire cesser la guérilla permanente des ennemis de l'école émancipatrice.

de dire que le fameux « pas de vagues ! » n'est pas ou n'est plus, si vous préférez, la logique de l'éducation nationale. Je l'ai dit dès les premiers jours de mon arrivée au ministère il y a trois ans et demi, et je l'ai démontré ensuite. Dans cette affaire, ce n'est pas le « pas de vagues ! » qui est en question. Bien sûr, il existe des problèmes,

de la défense sans faille des principes de la République. Oui, la peur doit changer de camp ! Oui, la foi ne saurait être au-dessus de la loi ! Mais si la parole a des vertus, elle a des faiblesses. La République doit éclairer, mais aussi protéger. Alors, commençons par modifier l'article 431-1 du code pénal. Je tiens une proposition de loi

Chacun ici a soutenu des gouvernements qui ont dû faire face au terrorisme. Cela doit tous- je m'adresse également au président Retailleau à cet instant -nous engager à l'humilité et à la responsabilité. Dans une période troublée et violente, il est d'autant plus nécessaire d'être clair sur les principes. Le premier principe est que la France est un État de droit, c'est-à-dire un pays où la norme s'applique et où l'arbitraire n'a pas sa place. Or, depuis vendredi, monsieur le Premier ministre, votre ministre de l'intérieur dit vouloir intimider et passer des messages, usant pour ce faire de pouvoirs qui trouveront rapidement leurs limites, et assume une forme d'arbitraire. Le garde des sceaux, tout d'abord discret- il est d'ailleurs absent aujourd'hui -, semble prêt à modifier la loi fondatrice de la liberté de la presse et de la liberté d'expression du 29 juillet 1881. Permettez-moi de vous rappeler les propos tenus par Robert Badinter, au lendemain de l'attentat contre : « Ce n'est pas par des lois et des juridictions d'exception qu'on défend la liberté contre ses ennemis. Ce serait là un piège que l'histoire a déjà tendu aux démocraties ; celles qui ont cédé n'y ont rien gagné en efficacité répressive, mais beaucoup ont perdu en termes de liberté et parfois d'honneur. » Monsieur le Premier ministre, dans cette période où le « en même temps » ne peut vous guider davantage, ma question est simple : entendez-vous écorner notre État de droit ou, au contraire, vous y référer toujours dans un face-à-face courageux avec les Français ?

pour la réplique. Je regrette, monsieur le ministre, que vous n'ayez pas affirmé votre attachement à l'État de droit.

Élu local, en trente ans, j'en ai vu et entendu des renoncements. J'ai aussi vu cette idéologie totalitaire gagner nos quartiers, encouragée par la lâcheté coupable de politiques et aussi de technocrates. On a fermé les yeux sur l'immigration massive liée au regroupement familial, sur la création de ghettos urbains, sur la dérive de ces quartiers gangrenés par la drogue, le communautarisme et l'islamisme. On a fermé les yeux sur les motivations réelles de certains migrants qui viennent pour porter la haine et le sang. On a fermé les yeux sur les coups de canif à la laïcité, les repas de substitution, les prières de rue, les couloirs dans les piscines, le port du voile dans l'espace public. Autant de coups de boutoir portés contre les fondements de notre République ministre, vous ne pouvez pas fermer les yeux, parce que l'horreur vous a sauté au visage, comme à nous tous d'ailleurs, parce qu'il s'est passé à Conflans la même chose qu'à Raqqa ou à Mossoul. Alors, que doit-on faire aujourd'hui ? Les Français ont compris qu'allumer des bougies et défiler dans la rue n'étaient pas un rempart contre cet ennemi qui veut imposer la charia au ventre mou de l'Occident. Les Français attendent de vous des actes forts : la mise en place d'une immigration choisie, et non pas imposée par des juges irresponsables ; l'expulsion des clandestins et des délinquants étrangers ; une application sans faille des règles de la laïcité ; la déchéance de nationalité contre tous ceux qui prennent les armes contre la mère patrie ; la reconquête, rue par rue, de toutes les zones de non-droit ; un soutien total à la police et, si nécessaire, le renfort de l'armée. Pour cela, il faut un exécutif déterminé et un Parlement respecté, car représentant légitime du peuple. Ils ne passeront pas », a déclaré le Président de la République. Le combat a donc enfin commencé chez nous- espérons-le ! Monsieur le Premier ministre, dites-nous avec quelles armes nous allons combattre et comment nous pouvons gagner cette guerre. Plus de renoncements, s'il vous plaît,

D'abord, vous faites un lien, que j'ai déjà entendu plusieurs fois, pas de la part de tous les représentants du groupe Les Républicains, mais de la part de quelques-uns, qui revient à dire : étranger égale islam, islam égale problème, problème égale terrorisme.

Nous ne contestons pas la pertinence de ce choix, qui relève presque du bon sens. Pour relocaliser, réindustrialiser et relancer, il faut effectivement alléger la fiscalité des entreprises.

On ne touche donc pas aux impôts de l'État, tels que la taxe sur les salaires, la C3S ou le forfait social. C'est toujours la même logique qui est à l'oeuvre, celle ayant déjà présidé à la suppression de la taxe d'habitation. La fiscalité locale est mise en coupe réglée. Le ministre des comptes publics nous a bien assuré que la baisse des impôts de production serait « compensée intégralement et de manière dynamique pour les collectivités ». mais cette politique sape encore une fois en profondeur le principe d'autonomie fiscale des communautés de communes ou d'agglomération. Lorsque l'on perçoit des dotations, aussi dynamiques soient-elles, on devient dépendant d'un État centralisateur. Supprimer les impôts locaux, c'est transformer les collectivités en simples guichets, car, sans fiscalité propre, on ne perçoit plus de retour sur investissement, et on n'a donc plus beaucoup de moyens n'a donc plus beaucoup de moyens ni de raisons de faire des efforts. Madame la ministre, on ne peut pas à la fois prétendre faire confiance aux territoires et aux élus locaux et poursuivre ainsi.

dans la population ! Comme vous le savez, les impôts de production baisseront de 10 milliards d'euros

mois, mais d'un virus dont la puissance contagieuse est connue mondialement depuis 1918 et pour lequel un vaccin existe depuis 1944.

pour éviter la rupture de stock en officines dès cette semaine, alors que nous entrons dans la période optimale pour se faire vacciner

j'ai apprécié le travail que nous avons pu mener ensemble l'année dernière, alors que vous étiez président du conseil départemental de la Vienne, sur la protection de l'enfance. La campagne de vaccination

devait s'adresser en priorité aux professionnels de santé et aux personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées et celles qui présentent un risque d'infection grave par la covid-19.

l'ensemble du système de soins, mais également protéger les patients avec lesquels ils sont en contact, notamment dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les

soient vaccinés, mais 75 %, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Compte tenu de l'anticipation d'une demande accrue cette année, nous avons fait le nécessaire pour mettre à disposition 30 % de doses supplémentaires par rapport aux 12 millions consommées lors de la précédente campagne.

à la constitution d'un stock d'État. Je peux donc vous assurer, monsieur le sénateur, que l'État fait tout pour protéger nos concitoyens de l'épidémie de grippe. La parole Je crains que nous ne devenions le pays de la pénurie : pénurie de médecins, pénurie de moyens dans les hôpitaux, pénurie de masques, pénurie de gel, pénurie de surblouses, pénurie de tests, pénurie de lits de réanimation, pénurie de doses de vaccin, pénurie d'anticipation, ce qui est encore plus grave plus grave ... L'impréparation est une faute, monsieur le secrétaire d'État. J'espère que nous allons nous mobiliser, les uns et les autres, pour qu'il y ait moins de pénuries et d'incurie dans ce pays. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

il a payé de sa vie la défense et l'enseignement de la liberté d'expression, de la laïcité, des valeurs de notre République. Il a payé de sa vie l'exercice d'un métier qui le passionnait, celui d'instruire et d'éduquer nos enfants. Avec le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, je m'associe évidemment à l'hommage qui lui est dû. Une de ses anciennes élèves indiquait hier : « Quand il entendait une remarque agressive contre moi en cours, il intervenait immédiatement pour me protéger. Je n'arrive pas à croire que personne n'ait réussi à le protéger, lui. » Nous partageons tous cette interrogation, nous disposons d'un arsenal juridique complet et de dispositions législatives et réglementaires spécifiques permettant, en théorie, aux pouvoirs administratif et judiciaire de prévenir la menace terroriste. Or, en l'espèce, à la suite des appels à la haine, de la campagne mensongère et diffamatoire et du cyberharcèlement dont ce professeur a été victime, et bien que des protagonistes soient fichés « S », nos services auraient conclu qu'il n'y avait pas de risque. Et pourtant, Samuel Paty n'est plus En 2014, le Parlement a introduit dans le code pénal les délits de provocation à la commission d'actes terroristes et d'apologie du terrorisme, et créé l'infraction d'entreprise individuelle de terrorisme. Dès lors, ces infractions peuvent donner lieu à l'emploi de techniques spéciales d'enquête prévues par le code de procédure pénale. En 2015, nous avons élargi et encadré les moyens d'action de nos services de renseignement. Malheureusement, nous savons, depuis les attentats survenus la même année, que cela ne garantit en rien le risque zéro. Toutefois, l'enchaînement des actes conduisant à l'assassinat de Samuel Paty illustre dramatiquement le manque de moyens consacrés à la mise en oeuvre des dispositions légales, moyens pourtant nécessaires pour réagir de manière adéquate aux signaux qui auraient dû alerter. Aussi, monsieur le ministre, au-delà des effets d'annonce d'hier du Président de la République et du Gouvernement, de quels moyens concrets, humains et financiers, les pouvoirs publics seront-ils dotés afin de prévenir plus efficacement la commission de tels actes terroristes ? La parole est

Madame la ministre, le 26 novembre 2019, avec mes collègues corapporteurs Frédérique Espagnac et Bernard Delcros, nous vous avons remis notre rapport portant sur l'avenir des ZRR.

un refus, et proposé une prorogation de seulement six mois, jugeant que vous auriez, en si peu de temps, la possibilité de réformer l'ensemble des critères de classement. Vous deviez également vous inspirer du travail sénatorial. Malheureusement, cette réforme n'a pas encore vu le jour, au point qu'aujourd'hui vous seriez prête, selon certaines informations, à proroger le système actuel jusqu'en 2022. Si cela est vrai, je m'en réjouis, mais je constate que le Sénat a de nouveau eu tort d'avoir raison trop tôt

peut-on parler d'un plan de relance, lequel contiendrait des mesures de relocalisation, alors que l'on s'apprête à réduire encore les ZRR, qui, comme on le sait, favorisent l'installation des entreprises dans les territoires les plus isolés ?

le demandaient les maires ruraux et le secrétaire d'État Joël Giraud, établir une géographie prioritaire de la ruralité plus ciblée.

commencé à le faire, notamment avec l'Insee, pour définir une nouvelle géographie de la ruralité dans les années qui viennent.

On connaît les réticences du Parlement, qui se demande si l'AFD n'a pas d'autres priorités que de prêter 250 millions d'euros à la Chine pour financer sa transition écologique. La semaine dernière, avec le concours du président Cambon, j'ai demandé au directeur général de l'AFD s'il n'était pas possible de redéployer ces prêts à la Chine vers le monde Indo-Pacifique,

Et de nous expliquer, geste circulaire à l'appui, que les Chinois achètent des obligations émises par l'AFD sur les marchés financiers, que cet argent retourne ensuite en Chine sous forme de prêts de l'AFD, une commission au passage ... au risque de servir la stratégie d'influence du régime communiste chinois à l'international. Cette situation de conflit d'intérêts est consternante. J'observe au quotidien les difficultés de nos entrepreneurs, qui se battent à l'international, et particulièrement en Afrique. Ils sont confrontés à des concurrents chinois utilisant des techniques commerciales interdites par notre droit. Ce conflit d'intérêts a fait réagir, en particulier, nos collègues d'outre-mer Nassimah Dindar, de La Réunion, ou Gérard Poadja, de Nouvelle-Calédonie. Celui-ci m'a alerté sur le prêt controversé de l'AFD à la Nouvelle-Calédonie, la lourdeur des réformes fiscales qu'il impose et les conditions opaques de sa conclusion. Selon lui, si l'influence de la Chine dans cet organisme prêteur était avérée, cela ne serait pas neutre pour l'avenir d'une partie du territoire français stratégique pour la France comme pour la Chine. Monsieur le ministre, la politique française d'aide au développement passe par l'AFD ; comment pouvez-vous garantir que cet organisme ne serve pas, malgré lui, d'autres intérêts que ceux de la France ? Quand le Parlement pourra-t-il disposer d'un rapport d'évaluation de la relation de l'AFD avec la Chine ? La parole

Nous agissons avec la Chine, sur ce point, pour lutter contre le dérèglement climatique. De surcroît, j'observe que cela présente des avantages pour les entreprises françaises, car l'intervention de l'AFD et de ses outils bancaires dans ce pays, sur ces sujets-là,

Pour vous, la barbarie ne serait qu'à nos portes, quand des gamins se font tirer dessus au Bataclan, quand des familles se font écraser à Nice, quand des passants se font poignarder, quand des profs sont décapités. La réalité, c'est que les barbares sont là, parmi nous, et qu'en plus nous n'avons plus de porte à fermer. Mes chers collègues, de droite comme de gauche, toutes les barrières, toutes les frontières. Ce que vous appelez timidement le « désordre migratoire », qui est, en réalité, une anarchie, une déferlante migratoire, vous en êtes tous responsables, à droite peut-être davantage, davantage, car c'est Nicolas Sarkozy qui a aboli la double peine ; c'est lui qui entretenait les meilleurs rapports avec le Qatar ; c'est sous sa présidence que l'immigration a battu des records. Mes chers collègues de droite, vos coups de menton d'aujourd'hui sont aussi indécents qu'inaudibles.

la politique d'immigration anarchique tue des Français, des terroristes d'importation tuent des innocents, mais, dans la classe politique, c'est le grand silence. Impossible pour vous d'avouer que la politique d'immigration, loin d'être une chance, est un véritable fléau. Il faut pourtant la stopper, car elle coûte trop de vies à la France Vous avez épuisé votre crédit communication, monsieur le ministre : il s'agit désormais d'agir pour sauver des vies. Malgré les insultes et les violences, le mouvement national auquel j'appartiens vous alerte inlassablement depuis des décennies.

Vous évoquez des attentats, tous horribles, tous ignobles,

sont allés en Syrie et en sont revenus pour commettre des attentats ignobles. Oui, il y a des étrangers radicalisés, mais éliminer les étrangers n'éliminera pas la radicalisation, monsieur le sénateur.

Il va être procédé, dans les conditions prévues par l'article 86 du règlement, au scrutin secret pour l'élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République. Ce scrutin se déroulera dans la salle des Conférences ; la séance ne sera pas suspendue durant les opérations de vote. J'invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité en se rendant aux deux bureaux de vote,

Je rappelle que la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être élu. Pour être valables, les bulletins ne peuvent comporter plus de six noms pour les juges titulaires et plus de six noms pour les suppléants. Le nom de chaque titulaire doit être obligatoirement assorti du nom de son suppléant. En conséquence, la radiation de l'un des deux noms, soit celui du titulaire, soit celui du suppléant, entraîne la nullité du vote pour l'autre. Une seule délégation de vote est admise par sénateur. Je remercie nos collègues Victoire Jasmin et Jacques Grosperrin, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin. Les juges titulaires et les juges suppléants à la Cour de justice de la République nouvellement élus seront immédiatement appelés à prêter serment devant le Sénat. Je déclare ouvert le scrutin pour l'élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République. Il sera clos dans une

3 voix pour, 25 voix contre -à la nomination de M. Thierry Coulhon à la présidence du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. J'informe le Sénat qu'ont été publiées des candidatures pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental et de la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ».

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, les Françaises et les Français qui ont atteint l'âge de la retraite s'endorment chaque soir sur une épargne de 5,4 milliards d'euros. Ce serait une excellente nouvelle pour leur pouvoir d'achat s'il ne s'avérait que, pour la plupart d'entre eux, cette épargne demeure invisible, ignorée, inconnue. 70 ans, le problème demeure : l'encours des contrats d'épargne retraite non liquidés s'élève à pas moins de 1,8 milliard d'euros. Je n'ignore pas que notre littérature est friande de ces héritages miraculeux, qui attisent toutes les convoitises c'est bien ce qui pousse le Tartuffe de Molière à conspirer dans la maison d'Orgon ; ce qui, à en croire Balzac, attire la bourgeoisie de Saumur auprès d'Eugénie Grandet ; ce qui explique enfin, chez Flaubert, la réussite sociale de Frédéric Moreau. Mais

Les milliards d'euros que représentent les encours des contrats d'épargne retraite supplémentaire non liquidés ne sont pas un pécule que des intrigants veulent s'arracher, mais bien au contraire une épargne que des hommes et des femmes ont construite par le travail, une épargne de sécurité dont des dispositifs ont toutefois effacé le souvenir. Le cynisme pourrait laisser penser que c'est une bonne affaire pour l'État, qui se retrouve à terme le propriétaire de tous ces contrats en déshérence. Tel n'est évidemment pas mon point de vue, ni celui du Gouvernement, ni celui des assemblées : cette épargne constituée par le travail doit revenir aux travailleurs ; cette épargne constituée en vue de la retraite doit être utilisée au moment de la retraite. L'État n'est ni Tartuffe, ni Félix Grandet, ni Frédéric Moreau : il est au contraire un garant, un régulateur, un facilitateur. Tous les assurés bénéficiaires d'une retraite supplémentaire doivent être clairement informés de ce que les assurances leur doivent. Cette démarche avait été amorcée dès 2014 pour les contrats d'assurance-vie et les comptes bancaires la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui permettra de lever les derniers obstacles en matière de contrats d'épargne retraite supplémentaire, pour lesquels l'information a toujours été difficile à obtenir, de la part tant des gestionnaires que des bénéficiaires. Les obstacles sont importants : non seulement ces contrats n'ont pas de terme, ce qui rend délicate la caractérisation de la déshérence, mais surtout le lien entre les gestionnaires et les bénéficiaires est souvent « distendu », pour reprendre l'expression du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). En effet,

proposition de loi a gagné en efficacité et en rigueur. Nous sommes aujourd'hui en mesure d'aboutir à des dispositions non seulement utiles, mais également consensuelles.

Je le dis très clairement : le Gouvernement y souscrit totalement. À l'article 1, qui constitue le coeur du dispositif, la commission a renforcé le dispositif d'information sur les contrats d'épargne retraite supplémentaire ; il transitera par le site internet La mesure consiste à s'appuyer sur ce site, qui centralise et consolide déjà les informations sur les droits à la retraite de chaque personne pour les régimes obligatoires, de base et complémentaires. Il s'agit d'y ajouter l'information relative aux droits acquis aux termes de contrats d'épargne supplémentaire. Ainsi, chaque personne qui se connectera à ce site aura une vision consolidée de l'ensemble de ses droits à la retraite, qu'ils soient acquis dans les régimes obligatoires, de base ou complémentaires, ou par des versements sur les contrats d'épargne retraite supplémentaire. C'est un dispositif particulièrement efficace de lutte contre la déshérence des contrats. Les échanges d'informations entre les gestionnaires des contrats de retraite et le groupement d'intérêt public (GIP) Union Retraite, qui gère le site Info Retraite, ont été précisés par la commission. En aval de la promulgation de la loi, une convention permettra de définir plus précisément les modalités d'échanges de données dans le cadre prévu, qui assure la protection des données personnelles. L'article 2 prévoyait que le nouveau service d'information qui est au coeur de cette proposition de loi fasse l'objet d'une campagne de communication. Autant l'obligation de transfert des données et la prise en charge financière des entreprises gestionnaires relèvent strictement de la loi, autant les dispositions prévoyant une campagne de communication peuvent être envisagées, me semble-t-il, à un niveau infralégislatif. La position de la commission nous convient donc totalement. En outre, la publicité du service est déjà prévue à l'article 1 et il est plus que probable que la mise en oeuvre de ce service bénéficie d'importantes retombées médiatiques qui contribueront également à son succès.

Le Gouvernement partage le constat des difficultés majeures posées par cette expérimentation. Dans ces conditions, le Gouvernement apporte tout son soutien à cette proposition de loi et souhaite qu'elle puisse être promulguée dans les meilleurs délais pour permettre une mise en oeuvre dispositif. Lutter contre la déshérence des produits financiers, c'est renforcer le pouvoir d'achat en apportant aux retraités un complément auquel ils ont droit c'est renforcer la qualité du contrat en défendant l'idée qu'il doit être honoré ; c'est enfin, tout simplement, renforcer la protection des citoyens en les aidant à se repérer dans des dispositifs qui peuvent souvent soit régulateur, garant et facilitateur : voilà ce que les Françaises et les Français sont en droit d'attendre de l'État. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à excuser Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales, qui se trouve temporairement éloignée de nos travaux. La proposition de loi que nous examinons vise à lutter contre la déshérence des contrats d'épargne retraite supplémentaire. Ces produits de capitalisation sont souscrits par des entreprises au profit de leurs salariés, ou volontairement par des individus, comme c'est souvent le cas pour les professions libérales. Ils sont destinés à compléter les pensions des régimes de retraite obligatoires à la cessation de l'activité professionnelle. Les prestations sont versées sous forme de rente viagère, même si une sortie en capital est possible dans certains cas. Le souscripteur peut liquider son contrat à l'âge où il le souhaite, et non pas nécessairement au moment de son départ à la retraite. Le risque de déshérence des contrats de retraite supplémentaire est bien identifié, notamment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Ces montants confirment que ni l'âge légal de la retraite ni l'âge effectif de départ ne sont celui de la liquidation du contrat de retraite supplémentaire, qui demeure un choix du souscripteur. Aussi les contrats non liquidés ne doivent-ils pas nécessairement être regardés comme en situation de déshérence. Celle-ci devient plus probable si aucune liquidation n'a été sollicitée à un âge avancé ; elle n'est cependant pas certaine.

4,5 % des cotisations, tous régimes confondus, obligatoires ou non, pour 2,4 % des prestations. Ce sont donc des produits encore marginaux dans la construction de la retraite.

s'éteindre au profit des nouveaux plans d'épargne retraite prévus par la loi Pacte. L'initiative du présent texte revient à notre collègue député Daniel Labaronne, qui a cherché à traduire la recommandation émise par le Comité consultatif du secteur financier en réponse aux constats faits par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité préserver l'intention de l'auteur du texte et le coeur du dispositif proposé. De nouvelles fonctionnalités seront donc bien mises en oeuvre par le GIP Union Retraite en vue de renforcer l'information des bénéficiaires de contrats d'épargne retraite supplémentaire. Grâce à ces nouvelles dispositions, l'assuré qui consultera le site Info Retraite au titre de ses droits à la retraite obligatoire verra désormais s'afficher également les éventuels contrats d'épargne retraite supplémentaire dont il est bénéficiaire. Le mécanisme proposé repose sur un répertoire créé à cet effet, dans lequel les gestionnaires de ces produits d'épargne retraite verseront des informations relatives aux contrats et à leurs souscripteurs. Le GIP Union Retraite sera chargé d'identifier les souscripteurs et de mettre à leur disposition, au moyen de son service en ligne, des informations sur les contrats détenus. La démarche constructive que nous avons retenue s'est notamment concrétisée dans le travail réalisé par la commission sur l'article 1 de la proposition de loi. Au nom de la clarté du dispositif, la commission a procédé au transfert au sein du code monétaire et financier Il nous semblait cohérent d'inscrire ces dispositions aux côtés des nouveaux plans d'épargne retraite et non au sein du code de la sécurité sociale, la retraite supplémentaire n'y ayant pas sa place. Nous avons également souhaité renforcer les distinctions entre retraites obligatoires et supplémentaires sur le site Info Retraite, en dissociant le relevé de situation sur les droits à la retraite obligatoire et en prévoyant des mentions informatives renforcées. Nous avons Nous avons surtout voulu garantir l'efficacité de ce dispositif sans pour autant remettre en cause la protection des données personnelles ni le droit au respect de la vie privée. La commission s'est ainsi attachée à encadrer les informations transmises par les gestionnaires au groupement

Il conviendra d'évaluer l'efficacité du schéma retenu dans ce texte et de déterminer si des données complémentaires seraient de nature à renforcer de manière substantielle ce dispositif. Notre commission a supprimé l'article 4, qui prévoyait une expérimentation visant à confier à des généalogistes la recherche des bénéficiaires de contrats placés à la Caisse des dépôts Ce dispositif expérimental nous a paru comporter des lacunes juridiques. Il nous par ailleurs semblé que sa mise en oeuvre conduirait à communiquer à ces acteurs des données personnelles et bancaires, ce que nous n'avons pas jugé souhaitable. En outre, il faut noter que la déshérence porte principalement sur de petites sommes et non sur de gros contrats, qui sont bien connus de leurs souscripteurs ; or un tel dispositif ne vise pas à résoudre un problème de masse sur des contrats peu rémunérateurs. Enfin, la Caisse des dépôts et consignations assure une mission d'information, et non de recherche de bénéficiaires, sur les contrats en déshérence dont les sommes lui sont transférées. La commission a bien veillé à ce que le dispositif fonctionne, comme elle a également tenu à ce que ce texte, qui vise à renforcer l'information des bénéficiaires de contrats d'épargne retraite supplémentaire, n'ouvre pas la porte à une grande confusion entre la retraite obligatoire et l'épargne retraite. Aussi a-t-elle émis des avis défavorables sur les amendements visant à revenir sur les clarifications et encadrements qu'elle a pu apporter. Le texte issu des travaux de la commission répond aux préoccupations et recommandations de l'ACPR. Équilibré, il permet la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif tout en garantissant sa finalité et son encadrement. Soucieuse de parvenir à un accord avec son homologue de l'Assemblée nationale, notre rapporteur a proposé une solution de compromis sur un point de divergence à l'article 1. 1. Sur son initiative, la commission a adopté ce matin un amendement levant l'interdiction de transmission au GIP de données financières sur les contrats. Ces informations devront se limiter au strict nécessaire. Considérant les derniers échanges, je suis optimiste sur le devenir de ce texte à l'Assemblée nationale. J'espère, comme nos collègues députés, que cette utile proposition de loi trouvera à s'appliquer rapidement.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous avons bien compris le sens de la proposition de loi relative à la déshérence des contrats d'épargne retraite supplémentaire. Insuffisamment avisés de l'épargne constituée en leur faveur, de nombreux assurés ont en effet pu délaisser leurs capitaux, qui demeurent en conséquence en déshérence au bilan des compagnies d'assurances. Cette proposition de loi instaure plusieurs garde-fous pour prévenir le phénomène de déshérence des contrats d'épargne retraite supplémentaire, en offrant une meilleure information aux assurés. Elle a pour objet d'inciter les gestionnaires à communiquer toutes les informations qu'ils possèdent sur leurs clients au GIP Union Retraite. Elle a aussi pour finalité la mise en place par le GIP d'une campagne de communication, afin d'aiguiller les retraités vers le site Info Retraite ; ceux-ci pourront ainsi vérifier s'ils sont ou non bénéficiaires d'un contrat d'assurance retraite supplémentaire. Enfin, elle tend à inciter les entreprises à informer leurs salariés qu'ils sont bénéficiaires d'un contrat d'épargne retraite supplémentaire. Il nous paraît évident que tout ce qui peut permettre aux personnes ayant souscrit un contrat de faire valoir leurs droits va dans le bon sens. Renforcer le droit à l'information de petits épargnants est une bonne chose. Cependant, il nous semble que beaucoup a déjà été fait sur le sujet. Il s'agit en effet ici de compléter les dispositions adoptées sous la majorité socialiste en 2014 et en 2016. L'enjeu était de taille : on recensait, en 2012, 1,8 million de comptes million de comptes inactifs, pour un encours de 1,6 milliard d'euros. Cette situation très insatisfaisante était notamment le fruit d'un environnement insuffisamment réglementé et contraignant. Les dispositions de ce qui deviendrait la loi Eckert du 13 juin 2014 ont ainsi plutôt fait l'unanimité : ce texte a notamment renforcé les obligations de recherche et d'information pesant sur les institutions financières proposant des contrats d'assurance-vie au profit des souscripteurs et des bénéficiaires de ces mêmes contrats.

l'épargne retraite soit constituée de contrats dont l'échéance ne peut être déterminée à l'avance complique en effet les choses. Les assureurs rencontrent également de nombreux obstacles pour retrouver les titulaires des contrats : ils n'ont souvent que les coordonnées des entreprises qui employaient les épargnants. La connaissance imparfaite par les épargnants des droits qu'ils ont pu constituer tout au long de leur carrière est aussi une source de difficultés. Pour résoudre ces problèmes, la loi Sapin II du 9 décembre 2016 impose aux assureurs qui proposent des contrats d'épargne retraite supplémentaire d'informer chaque année les assurés sur leurs droits. Cette loi dispose également que les assureurs doivent soumettre un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre de l'économie. Ce document doit indiquer le nombre et l'encours des contrats non liquidés, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour informer les adhérents. Malgré toutes ces dispositions, des problèmes demeurent. Cela amène à s'interroger sur les contrats dont il est question aujourd'hui : les contrats d'épargne retraite supplémentaire facultative relèvent en effet, pour la majeure partie d'entre eux, d'une logique de capitalisation

Ces dispositifs d'épargne retraite sont peu fiables : la preuve en est la nécessité de légiférer sans cesse pour leur permettre de fonctionner correctement. La présente proposition de loi a donc pour objet de corriger des difficultés inhérentes à un système de retraite facultatif qui dysfonctionne. C'est la raison pour laquelle je m'interroge sur l'intérêt du texte discuté aujourd'hui. Ne devrait-on pas plutôt se pencher sur la forme et le fond de ces contrats ? Nombre d'entre eux ne sont jamais réclamés et des sommes d'argent dormant ne profitent pas à ceux qui devraient en être les bénéficiaires. Dans le même temps, elles permettent de financer on ne sait quoi, on ne sait où. Pourquoi donc continuer à aménager le droit pour améliorer à la marge des produits financiers qui, de toute évidence, sont insatisfaisants ? Ne devrait-on pas plutôt choisir d'améliorer les régimes généraux, puisqu'il est question de financer les retraites ? C'est ce questionnement de fond qui nous conduit à douter de l'opportunité de cette proposition de loi et qui détermine le choix du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain de s'abstenir. La parole

La loi Eckert du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence était un premier pas en direction de la sécurisation des bénéficiaires et des ayants droit de ces contrats. Elle a permis de renforcer les obligations de recherche et d'information de ces derniers par les institutions. Pourtant, les contrats sans terme que sont les contrats d'épargne retraite supplémentaire ne sont pas couverts par ces dispositions ou le sont de façon partielle. Les difficultés à retrouver les ayants droit s'ajoutent à la méconnaissance par ces derniers de leurs droits. Malgré les avancées apportées par les lois Sapin II et Pacte, l'accès à l'information des bénéficiaires et des ayants droit de ces contrats demeure un angle mort législatif que cette proposition de loi prévoit utilement de combler. Elle s'appuie, pour cela, sur les recommandations formulées par le Comité consultatif du secteur financier, ainsi que sur les rapports de la Cour des comptes et de l'Autorité de contrôle prudentiel et qui se sont saisies du problème. L'ACPR estime le montant des liquidités ainsi bloquées inscrites au bilan des sociétés d'assurances à 13 milliards d'euros en 2018. Le risque de déshérence des contrats obligatoires est plus important les salariés contractants n'ayant pas toujours connaissance, en pratique, de l'existence de ces contrats supplémentaires, qui concernent pourtant 4,5 % des cotisations et 2,4 % des prestations, comme l'a rappelé Mme Catherine Procaccia, rapporteur du texte.

Le GIP Union Retraite disposera, à cette fin, de nouveaux répertoires centralisant les données des souscripteurs fournies par les gestionnaires du produit d'épargne retraite. La commission des affaires sociales a apporté des modifications au texte initial, en prévoyant notamment un retour d'informations du GIP vers les gestionnaires, tout en préservant la vie privée et la protection des données personnelles des contractants. Mme le rapporteur a jugé opportun de supprimer les articles 2 et 4, l'article 2 étant désormais satisfait par la nouvelle écriture de l'article 1, l'article 4 ne présentant pas de garanties juridiques suffisantes. Pourtant, l'idée de confier à des experts en généalogie la recherche des ayants droit nous paraissait intéressante. En libérant ces liquidités, l'adoption de cette proposition de loi contribuera à redonner du pouvoir d'achat aux retraités. Elle s'inscrit dans la lutte contre le non-recours au droit.

Il ne s'agit pas d'un texte anecdotique : ces dispositions concernent 13 millions de Français qui disposent d'un contrat d'épargne retraite complémentaire, ouvrant droit à une rente moyenne de 195 euros par mois. Ce ne sont pas des sommes

Dans le cadre des contrats d'épargne retraite sans terme, la liquidation ne s'effectuant qu'après demande de l'assuré, les situations de déshérence sont nombreuses, en particulier lorsque la multiplicité des employeurs tout au long d'une carrière entraîne une multiplicité des contrats. La présente proposition de loi s'attaque à la cause première de déshérence : le manque d'information des contractants et des ayants droit. Nous la soutenons.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire aura davantage un rôle de prévention qu'un effet sensible de résolution du stock de contrats L'importance des montants en déshérence soulignait un des points de fragilité de ce troisième étage de retraite par capitalisation appelé à se développer à la suite des réformes successives des retraites, qui conduisent à une baisse tendancielle des revenus des retraités du régime général et et complémentaire obligatoire, dans un mouvement de substitution plus que de complémentarité, que nous dénonçons par ailleurs. Il convenait donc de rétablir la confiance dans ces produits, dont une partie des bénéficiaires ne faisaient pas valoir leurs droits, faute d'information ou parce que les organismes gestionnaires avaient perdu leur trace, ce qui souligne le défaut de fiabilité du système par capitalisation. Le montant de 13 milliards d'euros d'encours en déshérence est souvent évoqué.

est loin des chiffres souvent évoqués, même s'il reste non négligeable. Le texte de la commission des affaires sociales reprend l'obligation faite aux gestionnaires de ces produits d'épargne de transférer régulièrement leurs informations au groupement d'intérêt public Union Retraite.

c'est l'objet de l'article 3 -, il nous semble que, pour favoriser la connaissance par les salariés des contrats de retraite supplémentaire détenus, l'information doit être donnée sur le reçu pour solde de tout compte, comme retenu par l'Assemblée nationale et recommandé par le Comité consultatif du secteur financier. En conclusion, nous ne pouvons que souscrire à des améliorations dans le recours aux droits conventionnels, nonobstant notre critique de la volonté de promouvoir ce type de produits d'épargne retraite par capitalisation et de l'affaiblissement de notre régime général et complémentaire obligatoire de retraite Nous pensons par ailleurs que ces fonds en déshérence devraient,, être versés au régime général des retraites, plutôt qu'au budget de l'État.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire que nous examinons cet après-midi a été adoptée à l'unanimité le 22 juin dernier à l'Assemblée nationale.

l'identification des assurés et de leurs ayants droit se révèle souvent difficile, les gestionnaires perdant parfois leur trace au gré des ruptures de contrat et des changements d'adresse. Plusieurs lois régissent pourtant les obligations des assureurs en termes d'information et de paiement de leurs clients s'agissant des contrats d'assurance-vie, et donc d'épargne retraite. ni la loi Eckert de 2014, ni la loi Sapin II de 2016, ni même la loi Pacte adoptée l'année dernière ne s'attaquent précisément au problème de la déshérence de ces contrats de retraite. texte apporte une première réponse, afin d'éviter que ce phénomène ne perdure. Il prévoit ainsi que les droits relatifs aux contrats de retraite supplémentaire soient mentionnés sur le portail Info Retraite, avec obligation pour les assureurs de transmettre annuellement au groupement d'intérêt public Union Retraite un relevé de situation pour chaque assuré. L'article 1 prévoit en outre que cette communication se fasse aux frais des assureurs une convention négociée. L'article 3 dispose par ailleurs que les entreprises informent, travers du solde de tout compte, leurs salariés s'ils sont bénéficiaires d'un contrat d'assurance retraite supplémentaire. Ce texte a été partiellement modifié par la commission des affaires sociales, qui a souhaité mieux encadrer les échanges d'informations prévus entre le GIP Union Retraite et les gestionnaires. Sans remettre en cause les apports de la commission, les membres du groupe RDPI ainsi que plusieurs de nos collègues proposent de revenir sur l'interdiction de transmission au GIP, par les gestionnaires, de données financières relatives aux contrats de retraite supplémentaire. Ces informations, à savoir le montant des contrats concernés, nous semblent en effet conditionner l'efficacité du dispositif. Les gestionnaires de produits et les associations de consommateurs se sont d'ailleurs accordés sur cette mesure dans le cadre des discussions menées du Comité consultatif du secteur financier. En outre, les craintes exprimées au regard de la protection des données ne nous semblent pas justifiées. Le décret d'application du présent article sera en effet examiné par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui vérifiera la proportionnalité entre la nature des données transmises et le caractère d'intérêt général de la mission. Dans la perspective d'un vote conforme par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants votera cette proposition de loi ainsi que l'amendement de compromis déposé ce matin par la rapporteure, Catherine Procaccia, dont nous saluons le travail de concertation. Nous regrettons qu'elle n'ait pu se joindre à nous aujourd'hui. Enfin,

Dans « retraite supplémentaire », il y a « retraite », et, bien que ce dispositif ne soit pas obligatoire par principe, il n'en demeure pas moins que son analyse pourrait relever d'une discussion générale sur notre système de retraites- ou plutôt nos systèmes de retraites. À cela s'ajoutent les amalgames entre retraite complémentaire, retraite supplémentaire, etc. Bref, les Français ne s'y retrouvent pas et, naturellement, les contrats en déshérence se multiplient. Comme le rappelait notre rapporteur, cette proposition de loi intervient après la publication de deux rapports, l'un de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en 2018, l'autre de la Cour des comptes, en 2019, faisant état de plusieurs milliards d'euros d'encours de contrats de retraite supplémentaire non liquidés. Si la déshérence Si la déshérence ne peut pas toujours être confirmée, certains bénéficiaires souhaitant attendre avant de liquider leurs droits, elle est une réalité dans de nombreux cas, notamment pour les retraités de plus de 70 ans, dont l'encours des contrats non liquidés représente tout de même 1,8 milliard d'euros. Autant d'argent dont nos aînés auraient pourtant grand besoin

ne traitait que des contrats assortis d'un terme explicite ou dont le bénéficiaire était décédé. Or les contrats de retraite supplémentaire n'ont pas de terme et prévoient en principe une sortie en rente viagère. Ils ne font donc pas l'objet de recherche de bénéficiaires et, si le décès de l'assuré reste inconnu de l'assureur, la créance n'est pas éteinte. Afin de pallier le manque d'information des assurés, notamment lorsqu'ils quittent leur entreprise, la proposition de loi crée une obligation, pour l'employeur, d'informer le salarié sur son contrat de retraite supplémentaire au moment du solde de tout compte. Elle prévoit surtout des échanges d'informations entre les assureurs et le GIP Union Retraite, qui alimente le site Info Retraite. Désormais, les Français qui s'y connecteront pourront avoir connaissance de l'ensemble des contrats de retraite souscrits à leur nom tout au long de leur carrière. Les amendements de notre rapporteur adoptés en commission apportent globalement des précisions utiles sur les informations transmises par les gestionnaires de contrats au GIP Union Retraite, afin que ne soient communiqués que les éléments indispensables, sur les informations présentées sur le site Info Retraite, afin de préciser que les contrats de retraite supplémentaire ne relèvent pas des régimes obligatoires, sur un retour d'informations du GIP vers les gestionnaires, pour qu'ils aient connaissance du succès ou non de l'identification du souscripteur. Toutes ces avancées sont bienvenues. Je regrette néanmoins la suppression de l'article 4, qui mettait en place une expérimentation visant à confier la recherche des bénéficiaires de contrats en déshérence à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de successions. Nous pourrions peut-être trouver un chemin permettant la recherche active des bénéficiaires, tout en garantissant la sécurité des données personnelles. C'est pourquoi j'ai cosigné l'amendement n° 6 de notre collègue Jocelyne Guidez. Toutefois,

texte. Dans l'attente d'une grande réforme des retraites, le groupe RDSE votera en faveur de cette proposition de loi, qui apporte une réponse à la problématique des contrats non liquidés. Rappelons que la retraite supplémentaire représente tout de même 4,5 % des cotisations, tous régimes confondus. Dans un contexte de crise sanitaire et économique, la perte de ces prestations constitue, pour les assurés, une aberration à laquelle il nous faut remédier. Espérons que l'adoption de cette proposition de loi permettra d'assurer à nos concitoyens un accès effectif à l'ensemble de leurs droits. La parole

près de 2,6 millions de retraités devaient compléter leur pension du régime obligatoire par un contrat de retraite complémentaire, soit 13,9 % de plus que l'année précédente.

Dans ce contexte, cette proposition de loi visant à améliorer l'information aussi bien des personnes actives que des retraités sur les contrats d'épargne retraite supplémentaire dont ils auraient perdu la trace représente une avancée, l'identité de ses réels bénéficiaires : est-ce que ce sont les salariés et les retraités, qui pourront véritablement récupérer plus facilement l'argent placé depuis des années, des années, ou les assureurs, dont l'obligation de rechercher les titulaires des contrats est transférée au groupement d'intérêt public Union Retraite ? En 2014, la société Allianz s'est vu infliger une amende de 50 millions d'euros pour avoir tardé à retrouver les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie

souscrits directement par les entreprises, pour lesquels les assurés n'ont pas eu de contact direct avec l'assureur. Lors des débats de 2013 sur la loi relative à la sécurisation de l'emploi, qui entérinait l'accord national interprofessionnel, notre groupe avait fortement critiqué la mise en place des complémentaires santé obligatoires dans les entreprises, pointant le manque d'information des salariés et le risque de réduction des prestations couvertes par la sécurité sociale. De plus, l'évolution de l'organisation du travail conduit bon nombre de salariés à changer souvent d'emploi, ce qui entraîne la signature de nouveaux contrats collectifs obligatoires et rend illisibles, pour ces « polyassurés », leurs droits à la retraite.

être le cas, faut-il rappeler que l'article 50 du projet de loi prévoyait que, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation du texte, la Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) continuerait à assurer la mission d'information des bénéficiaires de contrats de retraite supplémentaire.

je tiens à saluer la qualité du travail effectué par notre collègue rapporteur Catherine Procaccia. Les auteurs de cette proposition de loi constatent que certains épargnants sont insuffisamment informés sur l'épargne qu'ils ont constituée

En dépit d'importantes avancées permises par la loi Pacte, qui étend ces dispositions aux contrats sans terme, et par la loi Sapin II, visant à renforcer l'information des salariés sur les contrats de retraite supplémentaire, le phénomène de Ces nouvelles dispositions sont insuffisantes aux yeux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans son dernier rapport, elle démontre que, à la fin de 2016, « les contrats de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire ou facultative non liquidés passé l'âge de 62 ans représentent environ 10,6 milliards d'euros [ ...] et s'élèvent encore à 1,8 milliard d'euros pour les assurés âgés de plus de 70 ans Comme la Cour des comptes, qui a proposé différentes pistes de travail, le Comité consultatif du secteur financier s'est saisi de la question et a rendu un rapport en janvier dernier.

En effet, l'essentiel du dispositif repose sur la création d'une nouvelle fonctionnalité renforçant l'information de l'assuré

Il nous semble que ce dispositif répondra aux attentes des gestionnaires qu'aux recommandations de l'ACPR et de la Cour des comptes. Cependant, la formulation retenue à l'Assemblée nationale nécessitant d'être nuancée, la commission y a apporté les rectifications nécessaires. En effet, il ne s'agit pas tant de consacrer un droit nouveau à l'information que de tenter de renforcer l'accès à l'information pour les épargnants. Sur l'ensemble des points du texte, la commission des affaires sociales a apporté plusieurs correctifs bienvenus. Elle proposera d'ajuster encore le dispositif concernant la transmission au groupement par les gestionnaires de données financières sur les contrats de retraite supplémentaire. Toutefois, nous regrettons que ces dispositions ne concernent que le flux. On peut douter de l'efficacité du dispositif d'information

de vue. Dans la version du texte adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, un article 4 nouveau tendait à résoudre le problème du stock. Cependant, la rédaction proposée soulevant de réelles questions de conformité constitutionnelle, notre commission l'a supprimé.

Celle-ci pourrait être mise à contribution pour améliorer la prise en charge de leur éventuelle dépendance. Même si certaines données tendent à démontrer que les montants en déshérence par bénéficiaire sont relativement faibles, il n'en demeure pas moins que les intéressés doivent pouvoir être retrouvés. J'ajoute que ces près de 2 milliards d'euros seraient les bienvenus pour alimenter la relance de l'économie.

son rapport annuel de 2019, la Cour des comptes avait elle aussi alerté sur l'accélération du phénomène de déshérence, les stocks de contrats non liquidés augmentant avec l'ancienneté des contrats. La somme en jeu est importante.

retraite. Elle n'est pas juste, car, alors que les victimes de ce phénomène ont parfois versé des primes d'assurance toute leur vie, elles ne peuvent bénéficier des droits acquis. L'ampleur du phénomène et la crise sociale conjoncturelle doivent nous pousser à agir.

Pour ce faire, un répertoire sera créé, au sein duquel les gestionnaires de produits d'épargne retraite supplémentaire verseront des informations concernant les bénéficiaires des contrats. Le groupement indiquera ainsi à l'assuré, au travers du site Info retraite, l'existence du ou des produits souscrits à son nom. retraite individuel numérique, accessible le portail Info retraite, sera ainsi enrichi des informations sur les régimes de retraite supplémentaire. Les professionnels chargés de gérer les plans d'épargne retraite devront assurer la prise en charge de ce service en ligne.

un rapport qui révèle que la dématérialisation généralisée des services publics laisse trois Français sur cinq sur le bord de la route, tant les démarches administratives en ligne sont complexes.

À l'âge de 45 ans, Marguerite a eu l'occasion de s'installer à son compte et elle est devenue chef d'entreprise. Mais, au terme d'une vie de travail et à la veille d'une retraite bien méritée, notre pauvre Marguerite décède, victime d'un accident ... Commence alors un parcours du combattant pour Aristide, l'époux de Marguerite.

Mais comment faire ? Marguerite est passée par plusieurs entreprises, dont la plupart n'existent plus aujourd'hui. Dans sa vie, elle a changé trois fois de nom. En outre, en plus d'avoir souscrit des contrats sous différents noms, elle a cotisé auprès de plusieurs compagnies

L'assureur de la première société dans laquelle Marguerite a travaillé, il y a plus de trente ans, la connaît sous son nom de jeune fille, alors qu'elle a changé trois fois de nom par la suite. Établir l'historique des données est donc une difficulté très difficile à surmonter pour que pour les assureurs puissent remonter jusqu'au bénéficiaire et verser les prestations.

Une information complète et facilement accessible permettra en effet aux bénéficiaires de juger en toute connaissance de cause s'il leur est utile d'entreprendre des démarches. Ce partage d'informations sera par ailleurs encadré. Le décret d'application de l'article 1 sera examiné par la CNIL, qui vérifiera la proportionnalité entre la nature des données transmises et le caractère d'intérêt général de la mission.

Alors que la déshérence des contrats de retraite supplémentaire concerne un grand nombre de nos concitoyens et que l'encours du stock des contrats non liquidés atteint plus de 10 milliards d'euros,

Ces deux produits d'épargne peuvent être souscrits afin de compléter la retraite de base des bénéficiaires. Toutefois, il arrive que ces contrats ne soient pas liquidés. Les assureurs ont parfois des difficultés à retrouver les bénéficiaires, leurs héritiers ou encore les bénéficiaires désignés des contrats d'assurance-vie.

Néanmoins, la commission des affaires sociales a considéré que leurs dispositifs, tels qu'ils sont conçus, présentaient des lacunes juridiques. En effet, ils ne satisfont pas aux exigences constitutionnelles de précision, tant pour l'objet que pour la mise en oeuvre du dispositif d'expérimentation.

de conserver et de restituer les fonds sur demande. Elle ne peut donc pas déléguer. Ensuite, les organismes d'assurance sont déjà chargés de la mission de recherche des bénéficiaires et ils l'assument plutôt bien. Il n'apparaît donc pas nécessaire de dupliquer cette mission en la confiant à des cabinets privés, qui devront par ailleurs être rémunérés, d'autant que la proposition de loi va contribuer à résoudre dans une mesure significative le problème de la déshérence de l'épargne retraite. De surcroît, le fait de confier une même responsabilité à de multiples acteurs

Ont obtenu : Mme. Chantal Deseyne, titulaire, et M. Stéphane Le Rudulier, suppléant, 269 voix ; Mme Catherine Di Folco, titulaire, et Mme Brigitte Lherbier, suppléante, 269 voix

M. Teva Rohfritsch, titulaire, et M. Bernard Buis, suppléant, 269 voix. Ces candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, ils sont proclamés juges à la Cour de justice de la République. Mmes et MM. les juges titulaires et Mmes et MM. les juges suppléants à la Cour de justice de la République vont être appelés à prêter, devant le Sénat, le serment prévu par l'article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République. Je vais donner lecture de la formule du serment. Il sera procédé ensuite à l'appel nominal de Mmes et MM. les juges titulaires, puis à l'appel nominal de Mmes et MM. les juges suppléants. Je les prie de bien vouloir se lever à l'appel de leur nom et de répondre, en levant la main droite, par les mots : « Je le jure. » Voici la formule du serment

M. Teva Rohfritsch, juge titulaire, et M. Bernard Buis, juge suppléant, qui n'ont pu assister à la séance d'aujourd'hui, seront appelés ultérieurement à prêter serment devant le Sénat. Mme la secrétaire d'État, mes chers collègues, comme le président du Sénat l'a rappelé dans cet hémicycle lundi, la République a été attaquée vendredi dernier, à Conflans-Sainte-Honorine et à Éragny. Le terrorisme islamiste s'en est pris à l'un de ses serviteurs, Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie, assassiné dans des conditions odieuses pour avoir enseigné la liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté de caricaturer, pris pour cible pour avoir porté les valeurs de la République. La Nation lui rendra hommage dans quelques minutes dans la cour de la Sorbonne. Pour que nous puissions tous nous associer à cet hommage, je vous propose d'observer un instant de recueillement en la mémoire de Samuel Paty.